en moins entre 2012 et 2019 -, tandis que moins de 65 000 places de crèches étaient créées sur la même période et qu'un nombre important d'assistantes maternelles prenaient leur retraite. retraite. Cette politique a, en outre, eu l'inconvénient d'être très coûteuse pour les finances publiques, puisque les économies réalisées sur le congé parental se sont retrouvées neutralisées par les dépenses supplémentaires destinées à faire fonctionner les nouvelles places de crèches.

Je vous remercie,

notre point de vue n'a pas changé. La situation que vous visez est celle du paiement et du versement de la pension par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (CAF). Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un impayé de pension et il paraît normal que le parent débiteur donne son accord pour que le paiement de la pension soit effectué sous la forme d'une retenue sur ses prestations familiales. Cela n'empêche d'ailleurs pas les CAF de recouvrer des impayés de pension, en les récupérant sur des prestations auxquelles a droit le parent débiteur, et ce sans son accord. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement

En effet, environ 30 % des pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont de manière irrégulière, ce qui pose évidemment de nombreux problèmes, notamment pour les familles monoparentales. Concrètement, ce sont souvent des mères qui se retrouvent alors dans une situation de précarité financière importante. Je vous rappelle que 700 000 familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, soit un million d'enfants pauvres. L'an dernier, lors de

Dans ce cas et à la demande du parent créancier, l'Aripa est autorisée à transmettre des données relatives à l'adresse et à la solvabilité du débiteur pour faciliter les démarches du parent créancier qui souhaiterait recourir à un huissier de justice.

ce qui rend cette mention utile. Ensuite, vous proposez de préciser le montant de la pénalité en cas de non-transmission de ces informations après un délai d'un mois. La loi prévoit déjà un régime de sanctions pour non-transmission d'informations, le délai, le montant, la procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement étant fixés par décret. En effet, l'article D. 582-2 du code de la sécurité sociale définit déjà l'ensemble de ces éléments, dont les pénalités applicables. Enfin, la disposition, selon laquelle le directeur de la CAF informe le procureur de la République d'un refus manifeste, est déjà couverte par le droit commun figurant dans le code de procédure pénale. Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable.

façons de faire qui sont peu appréciées des parlementaires, et j'en comprends évidemment les raisons. La commission n'a pas eu l'occasion d'examiner cet amendement, mais je suis évidemment tout disposé à ce que nous en débattions ici. Il s'agit d'un amendement qui va dans le sens des familles et de la fluidité du système, puisqu'il vise à clarifier les modalités d'entrée en vigueur de l'avancement du versement de la prime de naissance. Vous savez que cette question du moment du versement fait l'objet de nombreux

le versement de cette prime avant la naissance, et non pas une fois que l'enfant est arrivé. Comme l'article 35 le prévoit dans sa rédaction actuelle, la réforme s'appliquera aux grossesses qui atteignent leur sixième mois en mars 2021, c'est-à-dire les grossesses qui ont débuté après le 1 octobre 2020, pour un premier versement le 5 avril 2021. La rédaction des dispositions d'entrée en vigueur de cet article pose une difficulté technique pour les grossesses qui atteindront leur septième, huitième et neuvième mois en mars 2021.

aux règles encadrant le service des prestations de l'assurance maladie. Il est notamment précisé que, s'agissant des décrets instituant ces dérogations, l'obligation de consultation préalable des caisses de sécurité sociale pour toute mesure ayant un impact sur leurs comptes est remplacée par une obligation d'information. Cet amendement tend à maintenir une obligation de consultation, tout en permettant d'en adapter les modalités. Il pose un problème à la fois sur la forme et sur le fond. D'une part, la rédaction proposée me semble un peu compliquée si on la lit attentivement. Si l'on peut réduire des délais, je ne sais pas ce que veut dire réduire des modalités de consultation. Par ailleurs, il est précisé que ces délais et modalités pourraient s'organiser sous forme dématérialisée, à condition que cela soit strictement nécessaire et proportionné, ce qui ne me semble pas non plus très clair. Enfin, il est fait mention de la situation d'état d'urgence, ce qui introduit une forme d'ambiguïté, car le dispositif dont nous parlons n'est pas limité aux situations d'état d'urgence. d'urgence. D'autre part, sur le fond, l'amendement mentionne la réduction des délais de consultation des caisses, mais ne fixe pas de délai minimal. Or une consultation n'a de sens que si les administrateurs des caisses sont réellement en mesure de se prononcer. Dans les situations d'urgence, il ne sera pas possible de laisser aux caisses un délai raisonnable, me semble-t-il.

Le Gouvernement souhaite toutefois profiter de cet article pour demander l'autorisation d'imposer, dans les mêmes conditions, des règles dérogatoires en matière de droit à l'indemnité complémentaire que verse l'employeur à ses salariés en cas d'arrêt maladie. En l'absence d'une telle possibilité, le Gouvernement a pris une ordonnance, le 25 mars dernier, qui doit arriver à échéance le 31 décembre prochain. Il s'agit là de dispositions du code du travail qui n'ont aucune incidence sur les dépenses de l'assurance maladie, et qui n'ont donc pas leur place en LFSS. Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de les censurer si nous les adoptions dans ce texte. D'ailleurs, le Gouvernement ne semble guère se faire d'illusions sur le sujet, puisqu'il a demandé, parallèlement à la discussion de ce texte, une habilitation à prolonger les mesures prises par ordonnance dans le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Gouvernement a donc la possibilité de maintenir les mesures prises pour répondre à l'urgence. Il pourra, le cas échéant, nous proposer un dispositif pérenne dans le cadre d'un véhicule législatif plus adapté. Les deux amendements suivants sont

Blanc qui avait déposé cet amendement. Il tenait à souligner qu'il y avait une forme d'insécurité juridique à laisser en l'état l'article 36, notamment parce que cela viendrait complexifier l'articulation des règles légales et des règles conventionnelles en créant un concours de normes. normes. L'application du principe de faveur conduit une même entreprise à verser à la fois le complément d'indemnisation prévu par les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail à une partie des salariés et le complément d'indemnisation conventionnel aux autres salariés. La gestion des arrêts de travail en serait particulièrement désorganisée. Quel est l'avis du Gouvernement ?

indissociables d'un revenu de remplacement garanti au salarié en cas d'arrêt. Il s'agit d'un dispositif global, qui articule les indemnités journalières et le complément employeur. Ce dernier n'est jamais versé seul : il vient nécessairement compléter les indemnités journalières de sécurité sociale. L'attribution d'un complément employeur aura ainsi un impact sur les dépenses d'assurance maladie, madame la rapporteure, dans la mesure, et toute la littérature économique sur les arrêts de travail le montre, où un niveau plus élevé d'indemnisation a des effets sur le nombre et sur les dépenses d'arrêt maladie. Les dérogations proposées au complément employeur sont essentielles pour indemniser suffisamment les salariés, mais aussi les inciter au respect de l'isolement, dans un objectif de protection de la santé publique. Nous l'avons bien vu au printemps, d'ailleurs, lorsque, du fait de la durée du confinement, le complément employeur s'est interrompu pour les parents en arrêt pour garde d'enfant ou de personne vulnérable, et que nous avons fait le choix de basculer sur l'activité partielle pour assurer un maintien de revenu et le respect des impératifs sanitaires. L'objectif du Gouvernement est donc de disposer d'un arsenal législatif le plus complet possible

est à Mme la rapporteure. Il s'agit d'un amendement visant à préciser les pouvoirs dérogatoires donnés au Gouvernement au titre de l'année 2021 en matière de couverture des frais de santé. Il semble en effet pertinent de prolonger les mesures prises depuis janvier 2020. Une disposition législative est nécessaire pour cela. Toutefois, il convient de préciser que cette dérogation au droit commun vise à répondre aux conséquences de l'épidémie de covid-19. soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Les dérogations sont liées, bien évidemment, au contexte sanitaire induit par l'épidémie de covid-19. Ainsi, l'intention du Gouvernement est bien de circonscrire la prolongation de ces dérogations à cette épidémie. Nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

en dépit des gestes barrières et des efforts demandés aux Français, l'épidémie de SARS-CoV-2 a probablement vocation à perdurer, avec une succession de phases de pic et de reflux. Il se pourrait par ailleurs que le virus ait, à terme, un comportement saisonnier, à l'instar de nombreux autres virus respiratoires. Ainsi, il paraît intéressant d'envisager de nouvelles initiatives dans le cadre de la stratégie de dépistage et de diagnostic, au regard de la cocirculation du SARS-CoV-2 et de certains virus responsables d'infections respiratoires, tels que la grippe et la bronchiolite. Comme le souligne la Haute Autorité de santé dans son avis en date du 15 octobre 2020, la détection des différents virus vise à diminuer le taux d'admission en hospitalisation pour les patients aux urgences, à organiser des mesures d'isolement appropriées et à mettre en place une prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale. Elle est donc au coeur de la lutte contre l'épidémie. Les tests multiplex permettent de détecter simultanément chez un patient la présence des virus responsables d'infections respiratoires hivernales et du SARS-CoV-2. Ces tests grippe-covid, développés par plusieurs laboratoires, devraient prochainement venir renforcer l'arsenal de lutte contre l'épidémie. Il conviendrait, face à l'ampleur et à la gravité de la crise sanitaire, d'envisager l'utilisation de ces tests, à titre expérimental, par les pharmaciens d'officine. Cette mesure contribuerait, d'une part, à désengorger les laboratoires, aujourd'hui surchargés, et, d'autre part, à améliorer significativement la couverture du territoire en matière de tests en période de cocirculation des virus. C'est l'objet du présent amendement que de permettre aux agences régionales de santé (ARS) d'autoriser cette expérimentation d'une durée d'un an et son financement par le fonds d'intervention régional. Il tend à prévoir que les conditions et modalités de déploiement de l'expérimentation soient définies par un décret, et que celle-ci fasse, à son terme, l'objet d'une évaluation remise au Parlement.

Les pharmaciens jouent d'ores et déjà un rôle dans l'accès aux tests de détection du SARS-CoV-2, avec le déploiement des tests antigénique. Ils proposent également des tests sérologiques sous la forme de Trod. Il serait en effet intéressant qu'ils contribuent de même à la diffusion des tests multiplex permettant de détecter simultanément le SARS-CoV-2 et les autres virus hivernaux à partir d'un même prélèvement, tests pour lesquels la Haute Autorité de santé a défini le 21 octobre des recommandations d'utilisation. Il serait utile que le secrétaire d'État, s'il le veut bien, nous précise la stratégie du Gouvernement dans leur déploiement. Dans l'attente, l'expérimentation proposée va dans le bon sens et s'inscrit en cohérence avec le rôle des pharmaciens. C'est un avis favorable de la commission.

concernant les recommandations pour l'utilisation et l'inscription au remboursement de tests de dépistage combinés des virus respiratoires hivernaux et du virus SARS-CoV-2. Afin de tirer les conséquences de cet avis, le ministère travaille travaille déjà, madame la rapporteure, à l'inscription aux nomenclatures de cet acte dans les indications recommandées quand elles sont réalisées en ambulatoire. C'est un travail qui est en cours. est en cours. Deuxième raison, les agences régionales de santé peuvent d'ores et déjà financer certains dispositifs innovants à titre expérimental sur le fonds d'intervention régional, sans que des dispositions législatives spécifiques soient nécessaires. Pour ces deux

au travers d'un fonds de l'assurance maladie. Cette allocation est à la charge, jusqu'à présent, de l'État. C'est la solidarité nationale qui assure le financement de cette allocation, qui fait office de minimum social, en complément des pensions d'invalidité. En parallèle de ce transfert, l'exécutif prévoit, par la voie réglementaire, une revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité, en relevant le plafond de ressources de 750 euros par mois à 800 euros par mois pour les allocations dues à compter du 1 avril 2021. Cette revalorisation est la bienvenue, puisque l'allocation supplémentaire d'invalidité n'a pas été réévaluée depuis une dizaine d'années, à la différence d'autres prestations, telles que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain se félicite de cette revalorisation par décret, mais ne souhaite pas entériner le transfert à l'assurance maladie d'une allocation qui a pour objet, non de compenser une invalidité, mais bien de la compléter, comme d'autres minima sociaux. Philosophiquement, il revient à l'État de conserver cette mission redistributive. Nous nous opposerons, d'une part, à ce transfert, et vous proposerons, d'autre part, tout à l'heure, un dispositif afin de lutter contre le non-recours à cette allocation supplémentaire d'invalidité.

l'amendement n° 178. L'article 37 transfère donc le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) à la CNAM, au seul motif que l'allocation est liée à la pension d'invalidité. Or l'ASI est aussi un minimum social, qui vise à compenser par la solidarité les limites des mécanismes assurantiels. Il y a donc une logique à ce que l'État la finance. La vraie question, qui fait l'objet d'une abondante littérature, est plutôt celle de l'articulation entre l'ASI et les minima sociaux, en particulier avec l'AAH, dont le plafond de ressources est plus élevé. Puisque cet article n'apporte aucun bénéfice aux assurés, il s'apparente à une débudgétisation ; il est donc proposé de le supprimer.

Dans la lignée d'autres mesures que nous avons déjà dénoncées, il s'agit là, pour notre groupe, d'un désengagement de l'État. Nous nous y opposons et souhaitons, comme vous, madame la rapporteure, supprimer cet article pour que la solidarité nationale continue de porter ce fonds, alors même qu'en raison des décisions de l'État la sécurité sociale connaît des connaît des déficits liés à ces désengagements.

alors que l'ASI est une allocation qui compense le handicap. Il s'agit également d'un minimum social, qui, à ce titre, doit relever des prérogatives de l'État, comme l'a dit Mme la rapporteure. Pour ces raisons, nous refusons également le désengagement de l'État et demandons la suppression de cet article

donc pas d'obstacle de principe à ce que cette allocation supplémentaire d'invalidité, qui relève de la solidarité nationale, soit financée par la sécurité sociale.

l'ASI complète, vous le savez, la pension d'invalidité. Elle obéit aux mêmes conditions médicales et administratives d'accès ; donc ce transfert va permettre un meilleur pilotage du risque invalidité en autorisant une vision unifiée de ces deux dépenses, qui sont profondément complémentaires.

pour les bénéficiaires de la pension d'invalidité. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ne font pas forcément valoir leurs droits à l'ASI par méconnaissance de ce dispositif et de leurs droits. Cet amendement vise à faire porter sur les caisses d'assurance maladie une obligation d'étude du droit à cette allocation et d'information aux assurés concernés.

; par méconnaissance du dispositif, on estime que de nombreux assurés ne font pas valoir leur droit à cette allocation. Ils doivent donc vivre avec des ressources très faibles, alors même qu'une prestation de solidarité devrait leur assurer un minimum social. Pour remédier à ce non-recours, plusieurs pistes techniques sont à envisager. Pour autant, gardons à l'esprit l'importance de l'humain dans l'accompagnement social. La présence de personnel sur le terrain, des assistantes sociales de secteur en nombre suffisant devraient permettent de résorber ce non-recours. Au-delà de la réponse humaine, nous pouvons envisager aussi une approche plus

une obligation d'étude systématique du droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité et d'information aux assurés concernés. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est particulièrement sensible à la problématique du non-recours aux prestations sociales. Sa résorption Sa résorption constitue à nos yeux une politique majeure de lutte contre la pauvreté et de réduction des risques sociaux. Dès lors, il va de soi que tout mécanisme ou dispositif qui participe d'une meilleure effectivité de l'accès aux droits doit être soutenu.

Rappelons que le coût social et de santé à moyen terme du non-recours est estimé bien supérieur à la dépense supplémentaire qu'induit à court terme un accès aux droits amélioré et renforcé. Nous pourrions d'ailleurs évaluer de la sorte les coûts évités.

stabilisateur automatique, car elles se traduisent en consommation immédiate et quasi intégrale : c'est ce qu'on appelle l'élasticité parfaite. Par cet amendement, nous nous inscrivons dans la poursuite de la politique de mobilisation des organismes sociaux contre le non-recours aux droits des personnes situation de pauvreté et de précarité. l'éligibilité à l'ASI des titulaires d'une pension d'invalidité. Le législateur a prévu une telle obligation d'information pour les potentiels bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette nouvelle obligation permettrait de limiter le non-recours aux droits.

nous allons y remédier dans les meilleurs délais. Pour autant, l'évaluation d'un droit à l'ASI nécessite de connaître l'ensemble des revenus du foyer, notamment des ressources qui sont aujourd'hui inconnues des organismes qui versent les pensions d'invalidité : revenus du capital, revenus de travailleur indépendant, ou encore pensions alimentaires.

par Mme Micouleau, vise à permettre de mieux évaluer l'impact psychologique de la crise sanitaire de la covid-19. L'insécurité, l'imprévisibilité, ainsi que les mesures restrictives prises dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis de nombreux mois ont un fort retentissement psychologique sur nos concitoyens. Depuis plusieurs années, différentes expérimentations sont menées afin de permettre le financement des consultations et des suivis assurés par des psychologues.

allocations familiales, RSA, aides au logement -ne sont accessibles qu'après un délai de carence correspondant à trois mois de résidence stable. Si cette règle se comprend parfaitement en temps normal, à l'heure actuelle, en revanche, elle nuit terriblement aux Français établis hors de France qui se voient contraints de rentrer en France. Du fait de la pandémie, ils sont des milliers à avoir perdu leur emploi ou leurs affaires : ils ont dû quitter en quelques semaines, voire quelques jours, leur pays de résidence. Or c'est précisément au moment de leur arrivée en France que ces Français ont besoin d'être aidés, d'autant qu'il s'agit d'individus dont les réseaux de sociabilité doivent être entièrement reconstitués.

de revenir vivre dans notre pays. C'est pourquoi il a d'ores et déjà été décidé, dans le cadre des mesures exceptionnelles, de suspendre le délai de carence de trois mois prévu pour l'accès à la protection universelle maladie des assurés n'exerçant pas d'activité professionnelle. Cette disposition, mise en oeuvre entre le 1 mars et le 1 juin, pourra être réintroduite par ordonnance en application de l'article 4 du projet de loi autorisant la prorogation de l'urgence sanitaire. sanitaire. Pour le droit aux prestations familiales et aux aides au logement, aucun délai de carence n'est prévu, sinon le délai d'un mois applicable à tous les demandeurs et pour toutes les prestations, en vertu de la règle générale d'une ouverture des droits le mois suivant celui où l'ensemble des conditions sont réunies. Les Français qui reviennent en France peuvent donc en bénéficier dès leur arrivée, à condition d'y résider ensuite de manière stable, c'est-à-dire au moins six mois sur une année.

la dépendance de la France, comme de toute l'Europe, dans le secteur du médicament nous ont fragilisés plus que jamais. Aujourd'hui, 80 % des principes actifs sont fabriqués hors de l'Union européenne. La mondialisation et la course aux dividendes démontrent une fois encore leurs effets néfastes. Il est donc urgent de penser à une Europe du médicament, si ce n'est à une Europe de la santé, et de relocaliser la fabrication des princepsen Europe.

Il est donc primordial de mettre en place un système de contrôle de l'efficacité de cette nouvelle mesure. La création d'un comité de suivi sous trois ans nous permettrait de tirer le bilan du nouveau système d'accès précoce et compassionnel et de proposer des évolutions du dispositif si l'on se devait se compte que celui-ci comporte des blocages résiduels et ne remplit pas les objectifs fixés.

de mise à disposition des médicaments au public dans l'attente de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Ce délai peut être particulièrement long ; il est de 500 jours dans le cadre du droit commun et atteint 700 jours pour certains médicaments spécifiques. Il est donc primordial de se donner les moyens d'adopter ce dispositif et d'en évaluer l'efficacité. On entre dans une période de grande innovation, notamment en cancérologie, avec les biomédicaments et les biomarqueurs. L'accès à ces médicaments à la pointe de l'innovation se fera selon

nous n'avons pas retenu les propositions visant à alourdir sans impact majeur le parcours des médicaments innovants, afin qu'ils parviennent le plus rapidement possible aux patients. Nous accompagnons avec vigilance la dichotomie actée entre l'accès précoce, d'une part, et l'accès compassionnel, d'autre part. Leurs logiques sont désormais clairement distinctes. Si le premier promeut avant tout l'effort de recherche de nos laboratoires, le second permet que des soins de dernier recours soient apportés à des patients dépourvus de traitement adapté. Enfin, nous ne souhaitons pas, à ce stade, toucher aux fondements du financement de l'accès dérogatoire. Rappelons que ce financement repose sur une couverture intégrale par l'assurance maladie du médicament dans sa phase d'accès innovant, ce qui en rend l'acquisition parfaitement neutre pour les établissements de santé qui le distribuent.

n° 209 rectifié ? Cet amendement pose un double problème. D'une part, la nouvelle condition qu'il pose à l'éligibilité d'un médicament sans autorisation de mise sur le marché à l'accès précoce semble redondante avec la condition immédiatement précédente de forte présomption d'efficacité et de sécurité au vu des résultats d'essais thérapeutiques. D'autre part, le caractère innovant d'un médicament doit absolument rester une condition nécessaire à son éligibilité à l'accès précoce. Sans cette condition, le régime juridique de l'accès précoce serait dangereusement voisin de celui de la prescription hors autorisation de mise sur le marché d'un médicament déjà existant, donc non innovant. Ces deux circuits de distribution et de prescription répondent à des objectifs bien distincts : le premier a pour vocation d'accompagner la recherche ; le second, de venir en aide, à titre principalement compassionnel, à des situations thérapeutiques individuelles sans solution. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable

sur le marché. Or l'attribution souvent très précoce de celle-ci par l'Agence européenne du médicament contraindrait le laboratoire à formuler une demande d'inscription au remboursement dans un délai assez bref après cette obtention, alors qu'il ne dispose souvent que de très peu de données sur les effets réels de la spécialité, ce qui serait susceptible d'orienter l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) vers un service médical rendu dégradé. Aussi cet amendement vise-t-il à permettre un dépassement de ce délai de trente jours. Quel est l'avis du Gouvernement ? Vous proposez,

Vous proposez, madame la rapporteure, que la HAS puisse accorder à l'entreprise qui bénéficie d'un accès précoce un délai supplémentaire pour déposer sa demande de remboursement de droit commun. L'article 38 prévoit en effet que le délai maximum de dépôt d'une telle telle demande est fixé à un mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. C'est ce même délai qui est actuellement applicable dans le dispositif d'autorisation temporaire d'utilisation. Il nous paraît important de rappeler l'objectif du dispositif de l'accès précoce : il est de permettre l'accès et la prise en charge de certains médicaments de manière anticipée et dérogatoire, c'est-à-dire souvent avant même

qui reste évidemment l'objectif final. Par ailleurs, votre proposition reviendrait à adapter le financement au cas par cas, alors que la réforme dont nous discutons met en place des modalités de prise en charge unifiées et prédéfinies pour l'ensemble des produits, de façon à donner aux industriels et aux payeurs de la visibilité et de la prévisibilité. Votre proposition nous semble ajouter de la complexité et soulever des questions en matière d'équité de traitement. Enfin, je me permettrai d'ajouter qu'à ce jour les laboratoires ayant bénéficié d'une ATU ont été en mesure de déposer une demande de remboursement dans le délai imparti.

Notre groupe souscrit à l'objectif de simplification et de raccourcissement des délais de mise à disposition des médicaments innovants dans le cadre de l'accès précoce mis en place par l'article 38. Afin de garantir effectivement cet accès plus rapide lorsque la mise en oeuvre du traitement ne peut être différée, il convient d'encadrer le délai de réponse de la HAS en le plafonnant à un mois. Cet amendement est issu d'un travail avec l'organisation

Je tiens à rappeler que l'attribution de l'accès précoce n'a aucun intérêt à être accomplie dans des délais raccourcis, contrairement à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables, pour laquelle le délai d'instruction par la HAS peut représenter un véritable enjeu, pour l'industriel comme pour les patients.

en cancérologie. La HAS et l'ANSM doivent pouvoir s'appuyer officiellement sur l'expertise de l'INCa en matière de recherche clinique de phase précoce, en particulier au travers de ses centres d'investigation spécialisés

l'avis de la commission ? L'INCa est surtout un organisme fédérateur des différents acteurs de la prise en charge du cancer en France- unissant notamment l'État, l'assurance maladie, les associations de patients, les fédérations hospitalières et la recherche -, ayant pour mission de se prononcer sur l'accompagnement des patients couramment suivis.

acteurs. Afin que cette transparence soit néanmoins complète, il est indispensable que la HAS motive ses décisions de refus d'autorisation d'accès précoce au marché. Cet effort de transparence est essentiel

Toutes les conditions d'octroi d'accès précoce sont précisées au niveau législatif : leur appréciation sera, bien sûr, justifiée par les deux agences. La précision que vous indiquez relève,

aux médicaments innovants, des données de suivi des patients traités. Il est important que ces données intègrent, outre la valeur thérapeutique et les effets indésirables du médicament, le critère de la qualité de vie du patient.

Vous proposez d'élargir, monsieur le sénateur, le dispositif dérogatoire d'accès compassionnel pour les médicaments qui font l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à un stade très précoce, en supprimant le caractère très précoce de cette recherche et en assouplissant l'engagement du laboratoire à déposer une demande d'accès précoce. La disposition que vous visez ici constitue une dérogation à l'accès compassionnel, qui s'inscrit pourtant dans une démarche d'anticipation de l'accès précoce. Puisqu'il existe des développements dans l'indication, il y a donc une volonté commerciale du laboratoire. Cependant, la demande émane d'un prescripteur, dès lors que le laboratoire doit constituer un dossier pour demander une AAP. En effet, ces médicaments ont vocation à être rendus accessibles aux patients en échec thérapeutique sans délais,

ils doivent l'être. Les médicaments n'étant pas disponibles, il faut qu'ils acceptent de les mettre à disposition. Il s'agit donc d'ouvrir l'accès précoce et l'accès compassionnel par rapport au cadre général

Cet amendement vise à intégrer l'INCa dans la procédure d'accès compassionnel aux médicaments innovants, au stade de l'instruction du dossier, lorsque le médicament concerné vise un usage en cancérologie. en cancérologie. La HAS et l'ANSM doivent pouvoir s'appuyer officiellement sur l'expertise de l'INCa en matière de recherche clinique de phase précoce, en particulier au travers de ses centres d'investigation spécialisés dans les essais précoces de nouveaux médicaments. Si, en pratique, cette consultation a lieu depuis quelques années, il convient toutefois de la formaliser afin qu'elle ne dépende pas seulement du bon vouloir des acteurs.

Il convient, en effet, de mieux encadrer le recueil des données, en introduisant le critère de la qualité de vie des patients pour l'accès compassionnel aux médicaments innovants. Quel est l'avis de la commission ? Pour

de lutte contre l'antibiorésistance. L'utilisation des phages est, à l'heure actuelle, très limitée par l'insuffisance d'offres résultant de problèmes industriels de fabrication

Compte tenu du faible risque que représentent les phages et de leur potentielle utilité en complément des traitements classiques dans certains cas d'infections particulièrement graves- les infections ostéo-articulaires, urinaires, pulmonaires et cutanées notamment -, cet amendement vise à alléger les contraintes d'accès au marché, spécialement pour les préparations à base de phages répondant à des standards de qualité minimale définis par voie réglementaire, en permettant leur utilisation même lorsque toutes les conditions d'accès à un usage compassionnel ne sont pas remplies.

de définir un encadrement du recours aux phages dans le cadre d'infections bactériennes complexes résistant aux antibiotiques. Cet encadrement devra assurer une coordination à l'échelon national afin d'orienter et de valider le recours aux bactériophages L'allégement des exigences que vous proposez pour les préparations à base de phages n'est cependant pas envisageable, car il s'agit de médicaments : à ce titre, ces préparations doivent répondre aux exigences de la réglementation

les antibiotiques ne sont pas du tout efficaces, en raison d'une antibiorésistance manifeste. Ces pauvres gens étaient handicapés, alors qu'un traitement exceptionnel à base de phages aurait permis d'obtenir des résultats.

qu'elle émane de services qui ne connaissent pas vraiment l'utilisation qui est faite des phages ni les équipes qui travaillent sur ce sujet et qui souhaitent que l'on aille plus loin.

est à Mme la rapporteure. L'article 38 prévoit de réserver à l'usage hospitalier les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce, y compris pour des spécialités qui faisaient déjà l'objet d'un circuit de distribution en ville. Cela pose un problème d'accessibilité du traitement pour les patients bénéficiant déjà de ces médicaments dans le cadre d'une AMM prise en charge dans le droit commun. Bien que ces cas restent exceptionnels, l'amendement vise à maintenir, dans le circuit de distribution de ville, les médicaments sous autorisation d'accès précoce faisant l'objet par ailleurs d'une AMM pour d'autres indications.

que vous souhaitez amender, lequel permet aux médicaments n'étant pas réservés à l'usage hospitalier d'être automatiquement inscrits sur la liste de rétrocession, dès lors qu'ils font l'objet d'une autorisation d'accès précoce ou d'un cadre de prescription compassionnelle, sans préjudice de l'existence éventuelle d'un autre circuit de délivrance du médicament, au titre d'une autre indication. pour effet non pas de remettre en cause le circuit de dispensation d'un médicament qui serait déjà disponible en ville au titre de l'indication de son AMM, mais de prévoir un circuit de rétrocession,

préciser que l'entreprise assurant l'exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées, tant dans le cadre de l'accès précoce que dans celui de l'accès

qu'il place l'entreprise consultée dans une position de juge et partie. En effet, l'article 38 prévoit que l'élaboration du programme d'utilisation thérapeutique se fait à la charge de l'exploitant.

dès lors que ces derniers feraient l'objet d'une autorisation d'accès précoce ou d'une autorisation d'accès compassionnel, au titre d'une extension d'indication.

Si une grande partie des objectifs peuvent être atteints, l'absence totale de visibilité sur les niveaux de remise que vont devoir reverser les exploitants ainsi que la possibilité que les grilles prévues soient fixées sans prendre en compte la réalité de leurs contraintes font peser un risque majeur sur l'ambition de cette refonte,

y compris françaises, notamment celles pour qui il s'agit du premier produit. Elles pourraient ne pas être en mesure d'aller au bout du développement

l'avis de la commission ? Jusqu'à présent, la couverture rétroactive par l'industriel de l'indemnité que lui avait consentie l'assurance maladie pour financer une ATU se faisait sur une projection de ventes futures sur trois ans, ce qui présentait de nombreux risques pour la prévisibilité financière des plus petits laboratoires.

L'application d'une majoration de remise sur l'indemnité d'accès dérogatoire pour l'industriel dans le cas où un délai de 180 jours serait dépassé entre le dépôt de demande de remboursement et l'inscription au remboursement pose un double problème. D'une part, ce délai de 180 jours a été défini pour s'imposer aux pouvoirs publics dans l'inscription au remboursement des médicaments de droit commun, sans être pour autant respecté du fait de délais de traitement particulièrement longs de la commission de transparence de la Haute Autorité Ces délais n'étant pas imputables à l'industriel, il paraît incohérent d'en faire un motif de majoration des remises dont il pourrait être redevable à l'issue de la phase d'accès précoce. D'autre part, cette disposition consacrerait incidemment dans la loi un délai dont la nature demeure réglementaire.

cette réforme est d'accompagner les spécialités bénéficiant d'une prise en charge dérogatoire vers une prise en charge de droit commun. En effet, le recul que nous avons désormais sur le dispositif actuel des ATU nous a permis d'observer que l'absence de mécanisme incitatif à la négociation engendrait, pour certains de ces médicaments, une inertie dans les négociations et un maintien non justifié de la prise en charge dérogatoire, alors que l'objectif est d'aller vers la prise en charge de droit commun. Le dispositif de modulation des remises que vous souhaitez supprimer est donc clé. Les acteurs en sont convenus durant les concertations que nous menons avec l'ensemble du secteur, puis, depuis quelque temps, dans le cadre de cette réforme structurelle.

issues de la directive européenne Transparence. En revanche, les modalités concrètes de calcul des 180 jours au-delà desquels l'application des majorations de remise sera possible seront précisées par décret en Conseil d'État.

définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, concernant l'autorisation d'accès précoce aux traitements. aux traitements. Avec ce dispositif, les risques seraient de voir non seulement le niveau des prix des médicaments fixé de façon arbitraire, sans prendre en considération le modèle économique permettant la mise sur le marché de telle ou telle molécule, mais aussi certaines entreprises renoncer à demander un accès précoce, empêcherait les patients de bénéficier d'une autre solution thérapeutique. Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l'État, confirmée au mois d'août dernier, et à éviter ainsi que, par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s'aggrave. L'amendement

L'augmentation de cette enveloppe dédiée aux médicaments innovants et coûteux est donc financée par ponction d'autres enveloppes consacrées aux soins plus courants. Les établissements de santé, en particulier les hôpitaux publics, autofinancent largement le coût de l'innovation pharmaceutique, alors qu'ils participent grandement à son évaluation à travers les essais cliniques. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer les remises reversées par les laboratoires de l'industrie pharmaceutique à l'assurance maladie dans la construction de l'Ondam établissements de santé l'année suivante, afin d'éviter un autofinancement par les hôpitaux publics de l'innovation pharmaceutique.

Compte tenu des deux modalités possibles de prise en charge par l'assurance maladie pour les accès compassionnels- indemnité maximale réclamée par l'exploitant ou base forfaitaire annuelle définie par arrêté ministériel -et de l'absence de critère régissant l'application de l'une plutôt que l'autre, l'amendement n° 186 vise à assurer le mode de financement par indemnité maximale maximale dans les cas d'autorisation d'accès compassionnel visant à déboucher sur une autorisation d'accès précoce, afin que les mécanismes de prise en charge puissent bénéficier d'une certaine continuité.

Étant donné la nature très spécifique de l'accès compassionnel, qui ne peut être confondue avec celle de l'accès précoce, cette dualité de financement me semble souhaitable, notamment pour éviter les effets d'aubaine. Plutôt que l'adoption de cet amendement, je demande son retrait et un ralliement aux amendements de la commission, qui flèchent le financement de l'accès compassionnel vers les modalités de celui de l'accès précoce, dans les cas où le premier est accordé en anticipation du second. L'amendement n° 31 rectifié

les dépenses liées aux médicaments innovants sont déjà intégrées dans l'Ondam hospitalier et ne figurent pas dans le budget des hôpitaux comme des charges supplémentaires. Les remises visées par l'amendement, qui interviennent à l'issue de la phase d'accès précoce de ces médicaments, viennent en déduction rétroactive des montants consentis par l'assurance maladie

prévoit pas de base forfaitaire pour l'accès précoce : un barème est fixé en fonction du chiffre d'affaires et les modalités seront prises par décret après concertation avec le secteur, lequel a déjà été entendu sur le principe

le dispositif d'accès très précoce constitue une sorte de porte d'entrée vers l'accès précoce, il ne vous aura pas échappé que l'encadrement de ce dispositif est plus proche de celui de l'accès compassionnel. Il ne nous semble donc pas pertinent de vouloir aligner les critères de prise en charge entre ces deux dispositifs. Par ailleurs, la durée dans ce dispositif très précoce avant bascule vers l'accès précoce sera très courte, du fait de l'engagement pris par le laboratoire de basculer vers l'accès précoce. Dès que le médicament basculera

l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) pour la prise en charge des dispositifs médicaux non-inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables et à élargir cet avis à la base forfaitaire annuelle pouvant servir de base à la prise en charge des autorisations d'accès compassionnel.

Aussi, il ne nous paraît pas pertinent de soumettre de nouveau à l'avis préalable de l'Uncam la décision des ministres fixant une base forfaitaire annuelle par patient pour un médicament bénéficiant d'une prise en charge compassionnelle, alors que cet avis a justement été supprimé pour la RTU, dispositif auquel l'accès compassionnel succède.

L'un des objectifs essentiels de la refonte des ATU et RTU prévue à l'article 38 est la réduction du délai de mise à disposition des médicaments au public, après obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Celui-ci peut être particulièrement long, de 500 jours dans le cadre du droit commun- et encore n'intègre-t-il pas les produits sous ATU - jusqu'à 700 jours pour certains médicaments spécifiques, alors que la procédure devrait se dérouler en 180 jours. Tel est le constat effectué en 2018 dans le rapport sénatorial d'information d'Yves Daudigny, Catherine Deroche et Véronique Guillotin, sur l'accès précoce à l'innovation en matière de produits de santé. Si notre groupe partage l'objectif et la démarche ambitieux des

déjà vraisemblablement l'objet d'un contrôle sourcilleux des autorités, des acteurs pharmaceutiques concernés, n'en doutons pas, et, bien entendu, du Parlement. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

d'amélioration de l'information des patients, mais aussi de recherche clinique et d'évaluation de l'efficacité des médicaments innovants. Dans cette il paraît essentiel qu'un nombre important de données puissent être collectées et stockées dans le Health Data Hub, tout particulièrement les données dites en vie réelle, c'est-à-dire les données générées à l'occasion des soins réalisés en routine sur un patient, qui reflètent la pratique courante. Complémentaires des données issues des essais cliniques qui participent à l'évaluation des médicaments et à la fixation de leurs prix, les données en vie réelle constituent une opportunité d'affiner l'évaluation de l'efficacité d'un produit. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à inclure dans le Health Data Hub

mais à modifier les finalités du système national des données de santé, le SNDS, et à intégrer les données de santé en vie réelle dans les évaluations de la Haute Autorité de santé. Toutefois, les finalités du SNDS permettent déjà déjà de mettre en oeuvre des analyses de données en vie réelle, car elles prévoient les recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé, ce qui intègre l'évaluation de l'efficacité en vie réelle des traitements.

de confier l'hébergement de ces données à Microsoft Azure, la branche de services en ligne du géant américain. Heureusement, dix-huit organisations et personnalités, dont le Syndicat national des journalistes, ont obtenu du Conseil d'État l'arrêt du transfert des données de santé française

des entreprises allemandes. Cette histoire un peu rocambolesque démontre la nécessité d'un grand service public des données de santé associant les expertises des soignants,

sont refaites parce que les informations ne sont pas forcément disponibles sur le territoire national pour les différentes personnes ressources qui en auraient besoin. C'est donc un vrai sujet. Les informations inhérentes à la santé des patients devraient

Dans son rapport de septembre 2020 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS pour il n'existe pas d'obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l'issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l'État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d'extension d'indication thérapeutique, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée permettant l'obtention d'un prix élevé, et obtenir par la suite des extensions d'indication à une population plus large sans que le prix change. Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d'extension d'indication thérapeutique. J'ajoute que cet amendement a été suggéré par Aides, Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, MSF Access Campaign, Oxfam et les l'avis de la commission ? Le dispositif de cet amendement prévoit un rythme obligatoire triennal de révision à la baisse du prix de tous les médicaments, sauf pour ceux dont l'amélioration du service médical rendu serait significative et dont le rythme de révision à la baisse serait lui quinquennal.

d'un effet sur le long terme, voire sur la vie entière, les thérapies géniques sont des traitements innovants dont les prix peuvent être élevés et dont le remboursement pèserait sur les comptes sociaux. Vu la nature et la durée de l'effet attendu, il n'est pas rare que les prix demandés par les laboratoires pharmaceutiques, fondés sur la valeur du traitement, dépassent le million d'euros Afin d'éviter les à-coups budgétaires les années où de nombreux patients seraient traités, de ne pas limiter l'accès à ces traitements à certains profils de patients uniquement et de faciliter le pilotage de cet impact budgétaire sur plusieurs années, l'assurance maladie a émis l'idée que les thérapies géniques puissent voir leur remboursement et leur paiement au laboratoire étalés sur plusieurs années. Cet amendement rend cette technique budgétaire possible et laisse à la Caisse nationale d'assurance maladie le soin de répercuter, en fonction de l'accord entre le laboratoire et le Comité économique

Cet amendement ne me paraît pas tout à fait servir l'objet qu'il décrit, dans la mesure où il prévoit d'étaler dans le temps le remboursement par l'assurance maladie des charges supportées par les établissements de santé pour l'acquisition de médicaments innovants : on en revient au au débat précédent. Ces charges font déjà l'objet d'une couverture intégrale lors de la phase précédant l'inscription au remboursement. C'est d'ailleurs cette couverture qui sert ensuite de base aux remises rétrospectivement calculées

qu'il convient, nous semble-t-il, d'analyser en profondeur avant de légiférer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par ailleurs, l'étalement du paiement ne doit pas occulter la première question à se poser,

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Le parcours de soins des Français change et se diversifie. Habituée à une médecine excessivement curative, hospitalo-centrée et fondée principalement sur le traitement médicamenteux, la société française voit poindre une nouvelle vision de la santé, plus préventive, englobant des activités paramédicales et complémentaires aux traitements- exemple le sport-santé, les comportements alimentaires vertueux, la méditation et les thérapies de gestion du stress ou des troubles de l'anxiété -donnant pleinement sa place au patient. Ce dernier verra d'ailleurs son rôle croître dans les années à venir, dans la mesure où la digitalisation du suivi médical renforcera le « retour patient » dans le dialogue entre professionnels de santé. Qu'il s'agisse d'anticiper des maladies chroniques ou de compléter leur traitement, de mieux préparer certains dépistages, comme celui du cancer du sein, et d'améliorer les soins de suite, d'accompagner le grand âge et d'atténuer des souffrances aujourd'hui en croissance chez les actifs, certes non invalidantes, mais pénalisantes dans la vie sociale- exemple le burn-out, la dépression, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, les allergies chroniques -, ces traitements plus ou moins récents occupent une place qui doit être reconnue par l'assurance maladie. Cette prise en compte semble d'autant plus nécessaire que les flux d'informations, de plus en plus nombreux et souvent contradictoires, instillent une confusion certaine parmi nos concitoyens. L'insertion des médecines complémentaires et de traitements non allopathiques au sein des nomenclatures de l'assurance maladie permettrait donc de mieux orienter les patients. Cet amendement tend donc à créer un organisme spécifiquement dédié à l'évaluation des médecines complémentaires, alternatives et homéopathiques, ainsi qu'à la fixation d'un taux de remboursement, afin de tenir compte des produits et des traitements adoptés par un nombre important de patients et présentant un apport médico-social reconnu. Mes chers collègues, il ne s'agit pas de rouvrir un débat, pourtant utile et demandé, mais de mieux piloter notre politique de prévention, en accompagnant l'évolution du parcours de soins

intervient souvent en complément, pour atténuer des effets secondaires de traitements plus ou moins lourds, comme alternative en cas d'intolérance ou d'hypersensibilité médicamenteuse, ou encore en association avec avec un traitement conventionnel sans interaction médicamenteuse. Aussi demandons-nous un rapport, avec un délai d'un an laissant le temps à la nouvelle situation de produire ses effets, afin de nous assurer que le déremboursement de l'homéopathie n'a pas pour conséquence une réduction de l'accès à la santé pour certains patients en raison des coûts supplémentaires impliqués par la décision de déremboursement ou un report vers des médicaments traditionnels répondant aux besoins des patients, mais en définitive plus coûteux pour l'assurance maladie.

Pierre Dharréville. Cette mission d'information a mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c'est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation. Faute d'une actualisation régulière de cette liste, certains dispositifs médicaux continuent d'être pris en charge par l'assurance maladie à des tarifs élevés d'exception, alors qu'ils sont devenus d'utilisation commune. Le ministre de la santé avait répondu qu'il s'agissait d'une décision que l'on ne pouvait inscrire sans évaluation

Cet amendement rejoint les préoccupations exprimées dans le rapport de Catherine Deroche, de Véronique Guillotin et de notre ancien collègue Yves Daudigny.

pour pouvoir être réintégré sans risque de déstabiliser les financements des établissements hospitaliers qui l'utilisent. C'est donc un sujet que vous connaissez bien, mais ce n'est pas une modification législative qui nous apparaît, en tout cas à ce stade, nécessaire. Je m'engage, au nom du ministre, à ce que les services du ministère chargés de tenir cette liste veillent à dynamiser sa gestion pour qu'elle soit réservée aux dispositifs innovants et onéreux, ce qui était effectivement l'objectif initial de sa création.

Annie Delmont-Koropoulis. Mes chers collègues, nous connaissons une période formidable : une période où la recherche médicale et pharmaceutique produit des progrès thérapeutiques considérables, si bien que de nombreux patients atteints de pathologies lourdes et rares ont pu avoir accès à des stratégies de soins qui n'auraient pu être envisagées il y a encore quelques années ; une période où, si nous connaissons une crise sanitaire considérable, nous savons pouvoir compter sur nos chercheurs pour parvenir à trouver une solution vaccinale dans les prochains mois. L'innovation thérapeutique est une chance qui doit être offerte à chaque patient lorsqu'elle peut lui être apportée, mais cette innovation coûte cher, très cher, si bien qu'elle bénéficie d'un système de financement spécifique dérogatoire. La prise en charge à l'hôpital des traitements présentant un caractère innovant est en effet conditionnée à leur inscription sur la liste en Cette liste permet un accès facilité à l'innovation, certes, mais elle écarte de fait le recours aux produits qui n'y sont pas inscrits. C'est notamment le cas des médicaments évalués avec un niveau d'amélioration du service médical rendu (ASMR) mineur, au niveau IV de la classification de la HAS. Cet état de fait représente, dans l'élaboration des stratégies thérapeutiques, une difficulté pour certains praticiens et patients ne pouvant avoir recours à ces produits dont l'ASMR est certes mineure, mais existante. Aussi, afin de s'adapter à la réalité de l'innovation et prévenir toute perte de chance pour les patients, cet amendement tend à déverrouiller l'accès à la liste en sus pour les médicaments évalués avec un niveau d'amélioration du service médical rendu classé IV. Quel l'avis de la commission ? La demande d'inscription sur la liste en sus est accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications thérapeutiques considérées : l'avis de la commission de transparence de la HAS, les prix pratiqués à l'étranger s'ils sont disponibles, les éléments d'impact financier pour l'assurance maladie, ainsi que le montant de l'indemnité maximale de l'autorisation temporaire d'utilisation, le cas échéant. L'amendement vise à permettre que l'inscription sur cette liste intervienne lorsque l'avis de la commission de transparence de la HAS identifie une ASMR de I à IV. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

inscrit sur la liste en sus ou les médicaments présentant un intérêt de santé publique, par exemple. Ceux qui ne sont pas concernés par les conditions précédemment mentionnées peuvent intégrer une expérimentation ouverte en octobre 2019 au titre de l'article 51. Cette expérimentation vise à faire évoluer les conditions d'utilisation et de prise en charge des traitements médicamenteux onéreux au sein des établissements de santé en abrogeant notamment le critère de l'ASMR comme condition d'entrée dans la liste en sus. Donc, à ce double titre, je considère que votre requête est déjà satisfaite, notamment dans le cadre de cette expérimentation dont il faut, par définition, attendre les résultats avant d'en tirer toutes les conséquences.

Annie Delmont-Koropoulis. Mes chers collègues, la révolution génomique offre de nouvelles perspectives pour la médecine tant prédictive que préventive. Le séquençage du génome humain peut aujourd'hui être réalisé en quelques heures, pour un coût moyen de 1 000 euros. La médecine génomique est un enjeu majeur de santé publique ; elle constitue une chance, pour les patients atteints de pathologies graves, de bénéficier à la fois d'une prise en charge personnalisée et de nouvelles thérapies ciblées. En 2018, la direction générale de l'offre de soins a mis en oeuvre le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) pour soutenir l'innovation en biologie médicale et anatomocytopathologie. Bien que cette nomenclature soit un outil pérenne de financement de l'innovation, il demeure que son enveloppe fermée n'est pas suffisante. En outre, celle-ci n'inclut pas, à ce jour, les actes liés à l'analyse génomique, ce qui n'encourage pas leur utilisation auprès des patients, les privant d'une prise en charge spécifique qui améliorerait considérablement leur qualité de vie. À titre d'exemple, les « tests compagnons », devenus indispensables dans la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein, ne sont pas financés, laissant les établissements décider s'ils supporteront ou non le risque financier,

par le biais d'un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, les possibilités de création d'une nouvelle enveloppe, attenante à celle du RIHN, et spécifique à la médecine génomique, afin d'accompagner le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. Quel

Cette approche globale nous semble en effet plus opportune qu'un découpage par sous-type d'actes. Enfin, le Gouvernement soutient et accompagne déjà, avec l'Inserm, le plan France médecine génomique, que vous connaissez